Mes chers collègues, je vous rappelle que le port du masque est obligatoire dans l'hémicycle, y compris pour les orateurs s'exprimant à la tribune, conformément à la décision de la conférence des présidents réunie le 1 décembre dernier. dernier. J'ajoute que le masque se porte sur le nez ! J'invite par ailleurs chacune et chacun à veiller au respect des gestes barrières. L'ordre du jour appelle l'examen de deux projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation de conventions internationales. Pour ces deux projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d'examen simplifié. Je vais donc les mettre successivement aux voix.

et le vote sur la deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs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

chère Céline Boulay-Espéronnier, mesdames, messieurs les sénateurs, nous voilà donc réunis ce matin pour achever le processus législatif de cette proposition de loi visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs. Disons-le, ce n'était pas gagné d'avance, notamment parce que certains acteurs y étaient opposés. Ce texte vient compléter et moderniser la régulation du secteur du livre autour de trois enjeux le soutien apporté à nos librairies et le rétablissement d'une juste concurrence sur le marché du livre ; l'amélioration de la relation contractuelle entre auteurs et éditeurs ; enfin, l'adaptation de la collecte des oeuvres numériques. proposition de loi très attendue vise à compléter utilement la politique volontariste menée par le Gouvernement depuis 2017 en faveur de l'ensemble de l'écosystème du livre. Je pense, bien sûr, aux crédits courants d'intervention dédiés à la politique du livre et de la lecture, aux 53 millions d'euros qui sont ou qui seront déployés en 2021 et en 2022 grâce au plan de relance afin de poursuivre la modernisation des librairies et des bibliothèques, de généraliser le dispositif « Jeunes en librairie » de renforcer les achats publics de livres, sans oublier, bien sûr, le succès formidable de la généralisation du pass Culture, véritable aubaine pour les librairies. La décision du Président de la République de faire de la lecture la grande cause nationale illustre encore un peu plus le soutien que l'État apporte ce secteur essentiel. Si l'accompagnement financier de l'État est indispensable pour permettre à la filière de faire face aux mutations structurelles qu'elle connaît, il était aussi nécessaire d'adapter notre arsenal législatif. C'est tout le sens de cette proposition de loi dont l'initiative revient à la sénatrice Laure Darcos, dont j'imagine l'émotion ce matin. Le Gouvernement, en particulier le ministère de la culture, a tout de suite soutenu ce texte qui permet de réaliser le souhait formulé par le Président de la République le 21 avril dernier à Nevers de retrouver un prix unique du livre en égalisant le prix de l'expédition, ainsi qu'en objectivant le coût de ce service pour les livres commandés sur internet et livrés chez soi. Ce texte prévoit un certain nombre de mesures permettant de moderniser et d'adapter notre loi de prix fixe, en renforçant notre régulation du prix de vente du livre. Cette régulation a été au coeur de nos débats. Un opérateur propose aujourd'hui systématiquement la livraison quasi gratuite des livres, quelle qu'en soit la quantité et quel que soit le montant d'achat, alors qu'aucun autre acteur ne parvient à proposer une telle aubaine au lecteur. Force est donc de constater que cette pratique commerciale constitue une nouvelle forme de concurrence par les prix qui ne permet plus à la loi sur le prix unique du livre de 1981 de produire son plein effet. Tout l'objet de l'article 1 texte est de rétablir l'effet de cette loi. La proposition de loi permet également de renforcer l'information du consommateur en clarifiant la distinction entre livres neufs et livres d'occasion dans la vente en ligne. en ligne. Nous devons également veiller, comme nous l'a recommandé le médiateur du livre, à resserrer la pratique des soldes de livres dans le cadre de ventes directement opérées par les éditeurs afin de ne pas fragiliser l'économie des libraires. Le principe d'équité qui sous-tend cette proposition de loi doit également guider la recherche de solutions pour ce qui concerne les relations entre un auteur et son éditeur. Ce texte offre, par ailleurs, une base législative à l'accord interprofessionnel signé par le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l'édition en 2017, relatif à l'encadrement des pratiques de la provision pour retour d'exemplaires invendus et de la compensation intertitres. Toutes ces mesures permettront d'améliorer l'équilibre et la transparence dans les relations entre les auteurs et les éditeurs. Enfin, cette proposition de loi apporte un complément très attendu au cadre du dépôt légal des oeuvres à l'ère numérique. Alors que nous terminons Alors que nous terminons l'examen de ce texte, je remercie très chaleureusement Laure Darcos et Céline Boulay-Espéronnier pour le travail que nous avons mené

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, c'est avec une pointe de nostalgie et le sentiment du devoir accompli que je me présente devant vous aujourd'hui pour achever le parcours de la proposition de loi de notre collègue Laure Darcos visant à améliorer l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs. Nostalgie, car ce fut un beau parcours, parfois tortueux, entre notre première réunion de commission le 2 juin, la large adoption en séance publique par le Sénat le 8 juin et par l'Assemblée nationale le 6 octobre, et enfin le recours à la procédure de législation en commission le 23 novembre dernier. À chacune de ces étapes, j'ai pu ressentir l'enthousiasme communicatif de Laure Darcos, certes, mais également du monde de l'édition, qui a puissamment soutenu le texte et nous regarde aujourd'hui. Car, ne nous y trompons pas : la proposition de loi que nous allons- je l'espère ! -adopter aujourd'hui, sous des aspects parfois techniques, constitue en réalité une vraie révolution, qui sera très rapidement ressentie par nos concitoyens, et portera la marque des travaux du Sénat.

Les Français ont marqué leur attachement à ces commerces, à ces lieux de vie et de culture uniques, dès la réouverture l'année dernière. La fragilité de leur situation ne doit cependant pas être sous-estimée, et il nous faudra certainement y revenir dans les années qui viennent. qu'il s'agit de « renforcer l'équité entre les acteurs ». L'équité renvoie naturellement aux très ambitieuses dispositions de l'article 1, qui bouleversent le modèle économique des plateformes, fait de livraisons gratuites destructrices pour le commerce de proximité. Je n'ignore Je n'ignore pas les débats qui nous ont agités sur cette question, et je dois avouer que ma réflexion a évolué durant nos travaux. Nous avons ainsi eu des échanges animés et passionnants avec la rapporteure pour avis, Martine Berthet, et avec la présidente de la commission des Bien entendu, c'est une forme de pari que nous tentons ici sur la responsabilité des lecteurs, mais également des libraires à proposer des solutions attractives à leurs clients. Le troisième et dernier élément du titre mentionne « la confiance entre les acteurs ». Le terme de « confiance » a d'ailleurs été ajouté par Laure Darcos lors de la première lecture au Sénat. C'est un mot important, qui rend justice au travail de négociation et de conviction qui a été mené sur l'article 3 de la proposition de loi, particulièrement technique, mais qui ne vise à rien d'autre qu'à créer les conditions d'un dialogue plus équilibré entre les éditeurs et les auteurs. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale- je salue la rapporteure Géraldine Bannier -ont très utilement amélioré le texte sans revenir sur ses dispositions essentielles. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous propose d'exprimer par un vote conforme sur ce texte notre confiance dans la capacité des différents acteurs de la chaîne du livre à se saisir rapidement et pleinement de ces dispositions audacieuses et novatrices.

le texte que nous examinons aujourd'hui vise à soutenir le secteur fragile de la vente de livres, constitué de 3 300 librairies indépendantes réparties sur notre territoire. Les dispositions proposées visent essentiellement à rétablir une certaine équité entre les acteurs traditionnels, les libraires et les nouveaux entrants, à savoir les plateformes de vente en ligne. Ces dernières, à travers les services de livraisons à domicile gratuits ou quasi gratuits, sont responsables d'une distorsion de concurrence avec les libraires, qui ne disposent pas des mêmes moyens. L'éviction des établissements physiques par les grandes plateformes au moyen de leurs politiques tarifaires agressives n'est pas soutenable. Le risque d'uniformisation des choix de lectures qui en découle n'est pas acceptable. Les librairies représentent, avec les bibliothèques de nos collectivités, les premiers lieux d'accès à la culture et aux savoirs. Qui n'est jamais entré dans une librairie avec un seul livre en tête, pour en ressortir, une heure après, les bras chargés de livres ? C'est vrai ! La diversité culturelle et la richesse de la production littéraire sont intimement liées aux choix que nous faisons aujourd'hui pour préserver le réseau de librairies indépendantes. Aussi ce texte dépasse-t-il de loin son objet. Il s'attache à préserver notre première industrie culturelle et l'ensemble de la chaîne du livre. La création, l'édition, la fabrication ou encore la commercialisation d'un ouvrage sont le résultat de nombreuses étapes faisant intervenir de multiples acteurs. Je tiens à remercier de nouveau l'auteure de la proposition de loi, notre excellente collègue Laure Darcos. Elle nous livre un texte, je l'ai dit en première lecture, consistant et ambitieux. Je ne peux également que me réjouir de la position de l'Assemblée nationale et de celle de Mme la ministre, Roselyne Bachelot. a amené le Sénat à recourir à la procédure de législation en commission pour achever rapidement l'examen de la proposition de loi et rendre possible sa promulgation avant la fin de l'année 2021. L'article 1 vise ainsi à améliorer les conditions de concurrence sur le marché de la vente de livres entre les librairies

Cette disposition novatrice fera l'objet d'un rapport du Gouvernement remis au Parlement dans un délai de deux ans afin d'en estimer les effets. Nous serons particulièrement attentifs aux conclusions de ce rapport. L'article 2 vise à instaurer la possibilité pour les collectivités d'attribuer des subventions aux petites librairies indépendantes, en complément du dispositif de soutien fiscal dont elles bénéficient déjà. Cette mesure est attendue Cette mesure est attendue par les libraires comme par les élus. L'article 3 tend à faire obligation à tout éditeur en cessation d'activité d'adresser un état des comptes à tous les auteurs sous contrat avec lui. C'est une mesure de bon sens. Elle correspond à une demande des auteurs. Nous la soutenons sans réserve. sans réserve. pour la possibilité ouverte aux auteurs et à des groupements d'auteurs de saisir le médiateur du livre. Il s'agit également d'une demande exprimée par les auteurs, que nous soutenons aussi sans réserve. Nos libraires tissent dans nos territoires un précieux maillage culturel et social. Les Français y tiennent beaucoup. Leur rôle est indispensable : je pense à leurs conseils, à leurs sélections. Tout cela joue un rôle prépondérant aussi bien en termes de mise en avant de la diversité éditoriale, d'aménagement du territoire et d'animation culturelle. Il est certain que le maintien et le développement des librairies indépendantes doivent constituer une des priorités de la politique du livre. La levée du gage par le Gouvernement lors de la première lecture au Sénat s'inscrit dans ce sens. Elle est un signal positif envoyé à tous les acteurs de la filière du livre que notre groupe salue. Pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, le groupe Les Indépendants-République et

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, il y a un an, quasiment jour pour jour, je déposais sur le bureau du Sénat la proposition de loi visant à améliorer l'économie du livre et à renforcer l'équité entre ses acteurs. Vous comprendrez mon émotion aujourd'hui, m'exprimant devant vous, alors que nous parvenons au terme de l'examen de ce texte, qui me tenait particulièrement à coeur. Permettez-moi tout d'abord de remercier le président de mon groupe, Bruno Retailleau, le président de la commission de la culture, Laurent Lafon, et le président du Sénat, Gérard Larcher, qui ont accepté que ma proposition de loi soit soumise à l'examen du Conseil d'État. Ma gratitude s'adresse aussi aux différents rapporteurs, nos collègues Céline Boulay-Espéronnier et Martine Berthet, ainsi que la députée Géraldine Bannier. Toutes les trois ont porté sur ce texte un regard bienveillant et ont contribué à en améliorer la portée et le contenu. Enfin, je ne saurais oublier le rôle décisif que vous-même avez joué, madame la ministre, avec vos équipes de la direction du livre et de la lecture. Sans votre soutien et sans votre conviction qu'il nous faut renforcer la politique du livre à l'ère du numérique, ce texte n'aurait pu être inscrit à l'ordre du jour du Parlement. Ma proposition de loi n'est pas née du hasard ou d'une subite impulsion privée : elle est le fruit d'une lente maturation et résulte des attentes progressivement exprimées par les professionnels du livre- auteurs, éditeurs ou distributeurs. Dans le secteur du livre, il ne peut y avoir d'acte de création sans une confiance durablement établie, sans perspective d'avenir à long terme. En affirmant ce besoin constant de transparence, j'ai à l'esprit ce qu'écrivait Voltaire à son amie Madame du Deffand, brillante femme de lettres : Pour faire un bon livre, il faut un temps prodigieux et la patience d'un saint. » Ma proposition de loi se veut régulatrice, en aucun cas répressive. Si elle était lourdement et inutilement normative, elle n'atteindrait pas son objectif. Car l'économie du livre est fragile, ne la brutalisons pas. Mon propos est de la conforter. La France, je tiens à le rappeler, bénéficie d'une importante diversité de commerces de vente au détail : 20 000 points de vente physiques, dont 3 300 librairies indépendantes, employant 15 000 collaborateurs. Ce réseau forme un ensemble unique en Europe et dans le monde, qui contribue à l'exception culturelle française. Or ce fragile équilibre est aujourd'hui menacé par la montée en puissance de la vente en ligne, dont la part de marché ne cesse d'augmenter. Il est aussi menacé par la politique commerciale prédatrice d'Amazon, qui utilise sa puissance économique pour mettre en tension tout le secteur français du livre, notamment en proposant un tarif de livraison imbattable : 1 centime d'euro sans minimum d'achat. Aucune librairie ne peut s'aligner sur un tel tarif sans mettre en péril son activité ! Voilà pourquoi s'imposait, selon moi, la nécessité de légiférer. Non pas pour empêcher Amazon de commercer- qui pourrait y prétendre ? -, mais pour établir des règles de saine concurrence et permettre aux libraires qui le souhaitent de se développer eux aussi sur le canal de la vente à distance. Certains ont brandi la menace d'une augmentation du prix du livre pour le lecteur. C'est faux, bien sûr, et d'ailleurs impossible : depuis la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, dite « loi Lang », le prix du livre est identique sur tout le territoire. Laissons à la mesure que je propose le temps de produire ses effets. Je tiens, en la matière, à saluer deux apports de l'Assemblée nationale. Le premier consiste à autoriser les détaillants à pratiquer la gratuité des frais de port lorsque la livraison n'a pas lieu au domicile de l'acheteur, mais a lieu dans une librairie. Il s'agit, d'une part, de ne pas pénaliser l'acte d'achat sur internet et, d'autre part, de favoriser des initiatives permettant le regroupement de libraires indépendants sur des plateformes de vente en ligne. Le second tient à la possibilité de réaliser un point d'étape dans un délai de deux ans suivant la publication de l'arrêté interministériel. Ma proposition de loi ne peut cependant se résumer à cette seule initiative qui, j'en ai conscience, a fait couler beaucoup d'encre et suscité des débats parfois passionnés. Car je présente aussi un encadrement plus large des pratiques contractuelles dans l'édition littéraire et musicale. Je propose diverses mesures qui seront favorables aux auteurs, notamment en matière de provision pour retour d'exemplaires invendus, de compensation des droits issus de l'exploitation de plusieurs livres ou encore en cas de cessation volontaire d'activité et de liquidation judiciaire de l'éditeur. Un mécanisme de référé judiciaire est par ailleurs introduit lorsque la résolution de certains litiges est caractérisée par l'urgence. Enfin, je ne voudrais pas conclure sans mentionner un point important de cette proposition de loi : l'adaptation des modalités du dépôt légal numérique, nécessaire pour préserver notre capacité à enrichir le patrimoine documentaire de la France. Le texte que je vous invite à adopter définitivement aujourd'hui a pour ambition de tracer l'avenir du livre, donc de la création, de la diffusion de la culture et de l'accès à la pensée. Ensemble, nous aurons fait oeuvre utile pour conforter la présence du livre au coeur même de nos territoires, pour lutter contre la dictature de l'algorithme et l'uniformisation des contenus. Ainsi sera préservée la diversité culturelle à laquelle nous sommes tant attachés. Je vous remercie de votre précieux soutien, car, selon la formule d'André Malraux dans son hommage à la Grèce, prononcé à Athènes en 1959, « La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert.

cette proposition de loi est le prolongement de la politique culturelle française, qui prend ses racines dans la loi Lang, laquelle a fêté dernièrement ses quarante ans. Une politique fondée sur une idée simple : le livre n'est pas un bien de consommation comme les autres et, par conséquent, son commerce doit obéir à certaines règles, avec notamment un prix unique. Ce texte vise à actualiser cette politique en prenant en compte une nouvelle réalité, celle des géants d'internet, en particulier Amazon. Nous sommes largement favorables à ce texte et je salue une nouvelle fois le travail remarquable de Laure Darcos pour sa rédaction et pour avoir tenu bon face aux pressions intenses du géant américain dont elle a fait état en commission. Au-delà des livres, derrière les prix bas, la simplicité, l'ergonomie, la rapidité de livraison et les références infinies, prenons quelques instants pour évoquer cette entreprise et les menaces que son modèle fait peser sur notre société. En 2020, Amazon c'est 60,64 millions de tonnes d'équivalent CO2 émis, soit une augmentation de 19 % par rapport à 2019. Ce niveau d'émissions de gaz à effet de serre est équivalent à celui d'Israël, de l'Autriche ou de la Grèce. Amazon, c'est également des millions de produits neufs détruits chaque année une enquête a montré que dans un seul entrepôt la firme pouvait détruire plus de six millions de produits par an. Un rapport de l'Inspection générale des finances alerte sur la non-facturation de la TVA par plusieurs vendeurs Amazon 98 % des vendeurs enregistrés sur les contrôlées ne sont pas immatriculés à la TVA en France. Telle est la réalité des prix cassés ! Sur le plan social, le tableau n'est pas plus reluisant avec une généralisation des emplois précaires, mal rémunérés, faisant largement appel aux horaires de nuit et sous la menace de licenciements abusifs. Pour un emploi créé chez Amazon, le commerce de proximité perdrait 2,2 emplois en France. À ce sujet, le texte que nous examinons aujourd'hui permet de réguler en partie la menace que l'entreprise fait peser sur les librairies indépendantes. En proposant un tarif de livraison à 1 centime d'euro, Amazon bénéficie d'une distorsion de concurrence qui met à mal le modèle économique des 4 000 librairies qui maillent notre pays. L'article 1 vise à y remédier en proposant l'instauration d'un tarif réglementé pour la livraison de livres, déterminé par décret. Cette proposition phare de la proposition de loi, bienvenue pour réguler ce marché de manière efficace, nous semble relever du bon sens. Mais il semblerait qu'Amazon ne l'entende pas de cette oreille. Notre collègue Laure Darcos a révélé en commission les négociations purement commerciales qu'a souhaité engager la plateforme avec le législateur. Je n'y reviendrai pas, mais je la remercie de la transparence dont elle a fait preuve en affichant en plein jour ce genre de méthode ! Nous voterons l'article 1 de cette loi puisqu'il constitue un caillou nécessaire dans la chaussure du géant, en espérant qu'il ne soit qu'une première étape vers une régulation plus importante des pratiques de cette firme. Autre mesure d'importance de ce texte, l'article 2 permet aux communes et à leurs groupements de délivrer des subventions à des librairies indépendantes en difficulté, comme c'est déjà possible pour le cinéma. Cette mesure permettrait ainsi le maintien d'un réseau dense, y compris dans nos zones rurales. Les articles 3, 4 et 5 visent à introduire plusieurs améliorations bienvenues aux relations entre les acteurs du secteur, par exemple en permettant aux auteurs de saisir, préalablement à une action en justice, le médiateur du livre. Mes chers collègues, le livre est un secteur essentiel, tous les acteurs l'ont montré durant la pandémie. Les librairies ont fait preuve de leur résilience durant cette crise en affichant des pertes pour 2020 de seulement 3 % alors que les prévisions les plus alarmistes des pertes de 15 %, voire de 20 %. Les Françaises et les Français ont témoigné de leur amour pour ces acteurs culturels en retournant dans les librairies à chaque déconfinement. La présente proposition de loi tend à reconnaître cette réalité et à permettre de soutenir encore davantage ce secteur. Elle vise aussi à mettre un frein à l'appétit sans limite d'une entreprise qui ne respecte rien ni personne, à commencer par la démocratie parlementaire.

Madame la présidente, madame la ministre de la culture et des archives, mes chers collègues, la proposition de loi dont nous débattons se place résolument dans le sillon tracé, il y a quarante ans, par la loi du 10 août 1981, qui a institué le prix unique du livre. à en prolonger la portée pour adapter ses dispositions aux évolutions économiques imposées par les plateformes numériques. Ce travail d'actualisation législatif avait déjà été entrepris par la loi du 8 juillet 2014

Il aura donc fallu attendre sept ans pour que le législateur réagisse et défende l'esprit de la loi de 1981. Analysons avec lucidité ce conflit dialectique du sabre et du bouclier et prenons collectivement conscience que l'objectif idéologique d'Amazon est d'abolir le prix unique du livre. Ce que conteste radicalement le Goliath de Seattle, c'est la capacité d'un État à organiser le marché par des règles qui s'opposent à sa volonté de toutes les anéantir. Soyons lucides, ce qui est en jeu par ce texte, c'est notre souveraineté nationale, c'est notre faculté de soumettre aux principes votés par le Parlement une entité monopolistique supranationale qui souhaiterait limiter l'action de l'État à ses seuls domaines régaliens. La liberté que prétend défendre Amazon est celle de la loi de la jungle, celle du renard lâché dans le poulailler. La commission des affaires économiques du Sénat considère qu'il faudrait que les poules aient des dents pour lui résister, c'est-à-dire qu'il serait nécessaire d'aider les libraires indépendants à affronter la concurrence d'Amazon sur son terrain de la vente en ligne. Je pense, avec Laure Darcos, la commission de la culture et Mme la ministre, qu'il est plus simple et plus efficace d'interdire à goupil d'occire les gallinacés sans défense. Car, tant que nous serons dans l'incapacité d'empêcher Amazon de se soustraire à l'impôt, nous ne pourrons protéger efficacement les libraires indépendants. Il nous a été expliqué que la fixation d'un prix minimal du port des livres augmenterait son prix et éloignerait de la lecture les populations rurales. La réalité du marché du livre n'est pas celle-là. Près de 45 % des achats de livres sont réalisés dans les grandes surfaces généralistes et les grandes surfaces spécialisées. L'approvisionnement des lecteurs de la ruralité se fait principalement par ces deux réseaux. Comme l'a bien mis en évidence la rapporteure, Céline Boulay-Espéronnier, dont je salue la qualité du travail, « l'achat de livres sur Amazon est surtout le fait de catégories aisées et urbaines Mais l'apport essentiel de la loi Darcos n'est pas là. Il est dans la reconnaissance, par son article 2, de la librairie indépendante comme établissement culturel d'intermédiation pour la défense et la promotion du livre et de la lecture. En cela, ces librairies agissent complémentairement avec les bibliothèques, dont nous discuterons du statut tout à l'heure, lors de l'examen de la proposition de loi de Sylvie Robert, par un très heureux hasard du calendrier. Cela a été dit, la loi Darcos offre aux collectivités la possibilité d'aider les librairies indépendantes, comme l'avait fait la loi Sueur pour les salles de cinéma. Le Conseil d'État, judicieusement consulté sur ce texte par le Sénat, explique la portée législative essentielle de cette disposition : « Les Les finalités en jeu sont la préservation de la diversité culturelle- en particulier sous l'angle de la résistance à l'uniformisation des contenus inhérente au modèle économique d'une grande plateforme [ ...] -, le maintien de l'accès de tous les citoyens à la culture [ ...] par le contact avec un libraire jouant son rôle d'éveil, de de conseil et d'animateur de la vie culturelle. » L'objectif de la loi Darcos est celui-ci : faire des 4 000 librairies indépendantes un réseau culturel de proximité au service du livre et de la lecture. Chez moi, à Bourg-la-Reine, mon libraire joint aux livres qu'il a envie de partager une petite note manuscrite par laquelle il exprime les raisons de son choix. Voilà ce qu'Amazon considère comme une concurrence déloyale, parce que ses algorithmes n'ajouteront jamais au livre ce supplément d'âme qui en fait des objets culturels si particuliers. Voilà pourquoi une plateforme ne remplacera jamais une librairie,

Si j'osais filer la métaphore, je dirais qu'un livre est aussi une porte par laquelle on fait entrer le savoir. Le livre n'est à l'évidence pas un produit comme un autre ; il est le socle de la civilisation. C'est sans doute ce qui explique le consensus qui s'est formé autour de la présente proposition de loi pour protéger ces passeurs de livres que sont les auteurs et les libraires. Ce consensus, je ne peux que le saluer au nom de mon groupe Union Centriste. Le phénomène est suffisamment rare pour être souligné. Cela a été rappelé, l'Assemblée nationale n'a apporté que de menues modifications au texte issu de nos travaux. Je n'y reviendrai donc pas, pour me concentrer sur ce qui constitue à nos yeux les principaux apports de la proposition de loi. En premier lieu, bien sûr, son article 1 interdit la gratuité de la livraison de livres afin de contrer ce qui a pu être analysé comme une concurrence déloyale faite par Amazon aux librairies traditionnelles. Il s'agit ni plus ni moins d'adapter la loi du prix unique du livre à l'apparition des plateformes pour en garantir l'effectivité. Une réforme qui s'inscrit dans la droite ligne des lois de 2011 sur le prix du livre numérique et de 2014 interdisant les rabais pour les livres vendus à distance. Mais, j'y insiste, il ne il ne s'agit pas d'édicter une loi anti-Amazon. Les plateformes sont des acteurs économiques importants qui sont inhérentes à notre modernité. À leur manière, elles peuvent aussi participer au désenclavement des territoires. En l'occurrence, il n'est question que d'équilibrer les conditions de marché entre acteurs, pas de céder aux sirènes démagogiques du « GAFA bashing second lieu, et dans le même esprit d'équité, les dispositions visant à équilibrer les rapports entre auteurs et éditeurs vont dans le bon sens, qu'elles portent sur l'information des auteurs quant à l'exploitation de leurs oeuvres, sur la provision pour retour d'exemplaires invendus ou sur la compensation intertitres. La possibilité ouverte pour les auteurs et leurs organisations de saisir le médiateur du livre est aussi de nature à apaiser les situations potentiellement conflictuelles. Ces dispositions reprennent l'accord de 2017. En les transposant, la démocratie parlementaire entérine et conforte le dialogue de la démocratie sociale. Mais la disposition qui me tient le plus à coeur est sans aucun doute l'article 2, qui permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d'attribuer des subventions aux librairies indépendantes, qu'elles soient labellisées ou non. Les élus locaux que nous sommes le savent tous bien : lorsque la librairie ferme dans un bourg, c'est une bonne part de sa vitalité qui s'éteint. Les librairies sont des points de vie cruciaux dans les territoires que l'on ne peut pas laisser mourir. L'aide instituée n'est pas disproportionnée puisqu'elle ne pourra pas dépasser 30 % du chiffre d'affaires. Elle ne pourra donc pas être mise en place en dépit de toute réalité économique. Elle permet ce que l'on pouvait déjà faire pour les théâtres, et ce que la loi Sueur a aussi autorisé pour les cinémas de quartier. Il n'y avait aucune raison que, dans ces conditions, n'existât pas à l'échelon national un dispositif fiscal équivalent pour les librairies. D'autant moins que cette aide a été mise en oeuvre de manière ponctuelle par quelques régions. En conclusion, il ne me reste plus qu'à féliciter Laure Darcos d'avoir porté ce texte avec détermination ainsi que notre rapporteure, Céline Boulay-Espéronnier, pour l'excellence de son travail, et le président de notre commission, Laurent Lafon, qui a oeuvré à l'accélération de son parcours législatif. Mais c'est aussi grâce à vous, madame la ministre, que ce texte a pu si vite prospérer. Merci d'avoir démontré à quel point un véritable dialogue entre le Gouvernement et le Parlement pouvait s'avérer fécond ! Très juste

que les sciences, les lettres et les arts sont une chose d'État, une chose que chaque nation produit en corps, que la patrie est chargée de provoquer, d'encourager et de récompenser. C'est bien l'esprit français qui a décidé de faire des livres des biens singuliers parmi les biens, et qui exprime cette volonté à travers l'exception culturelle. L'économie du livre ne saurait être exclusivement soumise à la loi du marché. La République française pouvait-elle en faire autrement ? Libres sont ceux qui s'émancipent par le savoir que renferment les livres. Égaux sont ceux qui par un même instrument accèdent à la même connaissance. Fraternels deviennent ceux qui ont dans leur poche une fenêtre sur le monde, fenêtre sur l'autre qui n'est alors plus inconnu. Fort de cette conviction, l'État a depuis quarante années oeuvré pour soutenir le secteur par le prix unique du livre, et l'interdiction des rabais de plus de 5 %. Néanmoins, l'économie du livre se trouve aujourd'hui La révolution numérique s'est traduite par un changement des habitudes, avec des conséquences telles que le développement des livres numériques ou l'essor de l'achat de livres en ligne. Malgré un regain d'intérêt pour la lecture dans la période récente, l'économie du livre demeure un secteur fragile. Les librairies affichent ainsi une rentabilité nette parmi les plus faibles des branches du commerce, comme a pu le souligner l'auteure de la proposition de loi, Laure Darcos. L'enjeu est de moderniser et de sécuriser toute la chaîne du livre, allant de l'auteur au lecteur. La présente proposition de loi pose l'interdiction de la gratuité de la livraison du livre. Cette mesure est indispensable si l'on veut enrayer la concurrence inéquitable qui persiste entre grands acteurs de la vente en ligne et librairies physiques. On se voit proposer des livraisons à 1 centime, mais à quel prix d'un point de vue social et environnemental ? Il convient de revenir à un modèle réaliste et soutenable. Le texte apporte également une clarification bienvenue en imposant d'afficher de manière distincte sur tout support l'offre de livres neufs et l'offre de livres d'occasion. Cela devrait permettre d'éviter toute confusion sur l'application du principe d'unicité du prix du livre. Sur notre territoire, on compte 4 000 librairies indépendantes qui représentent 15 000 emplois. Leur part de marché régresse depuis le milieu des années 2000. Aussi, le dispositif proposé par ce texte est, encore une fois, bienvenu : il permet aux communes et à leurs groupements, après conventionnement, d'octroyer des subventions aux librairies et autres détaillants. À cette aide s'ajoutera le coup de pouce apporté par le pass Culture, qui, je le rappelle, peut être utilisé pour acheter des livres en librairie, mais pas pour passer des commandes en ligne. L'intitulé de la proposition de loi nous le dit : il s'agit de conforter l'économie du livre, mais aussi de renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs. Un rééquilibrage est à opérer dans les relations entre les éditeurs et les auteurs du livre imprimé et de la musique. Sur ce point, les avancées sont cruciales. Le texte consacre l'accord conclu entre le Conseil permanent des écrivains (CPE) et le Syndicat national de l'édition (SNE) en 2017. Il pose l'interdiction par principe de la compensation intertitres et encadre la pratique de provisions pour retours d'exemplaires invendus. Je salue cette réaction au constat de précarisation et de fragilité croissante des auteurs : on le sait, 8 % seulement d'entre eux perçoivent des revenus artistiques supérieurs au SMIC. Ne pas agir face à cette fragilisation serait se résigner à un appauvrissement du paysage littéraire français, ce que nous ne pouvons, à la commission de la culture, évidemment pas tolérer. Autre point, la saisine du médiateur du livre est étendue aux auteurs et à leurs organismes de défense. Le médiateur peut formuler des préconisations aux pouvoirs publics ; l'intérêt est aussi que les auteurs prennent part à la discussion et à la réflexion. Enfin, le texte prévoit d'adapter le cadre législatif du dépôt légal des oeuvres à l'ère numérique. Les contenus des services de communication au public en ligne établis en France font désormais l'objet d'une obligation de dépôt légal. Créé en 1537, le dépôt légal fait actuellement entrer dans les collections nationales un exemplaire de toute la production éditoriale française, qu'elle soit écrite, sonore, graphique, cinématographique ou audiovisuelle, sous forme physique comme numérique. C'est donc un élément essentiel de notre mémoire culturelle collective. Je tiens à saluer le travail de notre collègue Laure Darcos, dont le texte répond à un besoin profond que les deux chambres, comme le Gouvernement, ont su reconnaître.

Nous ne pouvons que nous réjouir de cet aboutissement, qui est l'illustration du travail collectif que vous avez mené en amont avec les professionnels. Le consensus autour de la proposition de loi témoigne, bien sûr, de sa nécessité et de son importance pour la filière du livre qui attendait des ajustements structurels. aussi de la place qu'elle occupera au sein de l'édifice législatif relatif au livre, s'inscrivant dans la tradition des textes fondateurs pour la protection des acteurs et pour la protection de la diversité culturelle et littéraire. proposition de loi était devenue impérieuse au regard des pratiques développées par les plateformes en ligne- et en particulier une, qui, en plus de la remise autorisée de 5 % sur le prix du livre, rendait gratuite la livraison. Ainsi, cette plateforme tirait de sa position dominante un avantage concurrentiel décisif face aux librairies traditionnelles, menaçant par là même leur pérennité et fragilisant le maillage territorial de notre réseau de libraires, auquel nous tenons tous. proposition de loi entre dans une problématique plus large, très contemporaine, à savoir la régulation des plateformes numériques, et singulièrement des Gafam. Si, au niveau européen, sont actuellement discutés le (DSA) et le (DMA), le Sénat a d'ores et déjà été moteur en matière de régulation, en étant notamment à l'origine de la création d'un droit voisin pour les éditeurs de presse. Le présent texte, en interdisant la gratuité des frais de port pour un livre commandé sur internet, sauf dans le cas d'une opération « » effectuée en librairie, constitue ainsi un nouvel instrument sectoriel ayant vocation à étoffer notre arsenal réglementaire. il s'agit d'une mesure d'équité salutaire dont il conviendra de surveiller l'application. En ce sens, le rapport d'évaluation introduit à l'Assemblée nationale est bienvenu, afin de s'assurer que les plateformes ne contourneront pas l'esprit de la loi. Il s'agit également d'une mesure favorable à la sauvegarde de l'environnement puisque nous pouvons espérer une diminution des livraisons et, partant, des flux de transport. Naturellement, le Sénat, en tant que représentant des collectivités territoriales, ne pouvait que souscrire à l'objectif de l'article 2, qui vise à permettre aux communes et intercommunalités de subventionner leurs librairies indépendantes, sous certaines conditions. que ce dispositif fait écho à la loi de 1992 de notre collègue Jean-Pierre Sueur concernant le subventionnement partiel des cinémas, il s'avère un formidable levier pour préserver et dynamiser l'attractivité des centres-bourgs et des centres-villes. Cet attachement des Français à leurs librairies de proximité, considérées comme des commerces structurants, a été particulièrement visible depuis la pandémie de covid-19. Rappelons qu'au tout début de l'année 2021, 85 % des personnes interrogées

Enfin, dans un contexte où la majorité des artistes-auteurs sortent ébranlés de la crise sanitaire, le rééquilibrage de la relation contractuelle entre éditeurs et auteurs d'oeuvres écrites et musicales se révèle opportun, comme le démontrait déjà le rapport Racine de 2020. C'est pourquoi la plus grande transparence recherchée par l'article 3, au travers de la reddition systématique et complète des comptes en cas de cessation d'activité par l'éditeur par exemple, est un moyen idoine d'y parvenir. D'ailleurs, dans les prochains mois, je crois que nous devrons continuer à avancer sur la question de la protection des artistes-auteurs et à nous interroger sérieusement sur les carences de notre modèle de rémunération des créateurs à l'ère numérique. Si des avancées ont eu lieu ces dernières années, nous ne pouvons nous satisfaire : du non-respect du droit d'auteur sur et par les plateformes, bien que des progrès aient été effectués, car la loi doit s'appliquer ; du déséquilibre dans la relation contractuelle entre les plateformes numériques créatives et les artistes-auteurs, sanctionnant en particulier les jeunes artistes et les émergents ; et enfin de la captation, par les intermédiaires numériques, d'une part disproportionnée de la valeur créée par les artistes. C'est un enjeu culturel de premier ordre pour la France et l'Europe, qui appellera la réaffirmation de certains principes- toute oeuvre exploitée doit être rétribuée à sa juste valeur -et qui nécessitera l'adaptation de nos mécanismes aux pratiques des acteurs numériques, comme cette proposition de loi s'y est attelée pour le secteur du livre. livre. Sans surprise, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera ce texte. À titre personnel, je vous renouvelle, chère Laure Darcos, toutes mes félicitations et tous mes remerciements pour cet excellent texte.

mes chers collègues, la crise sanitaire a révélé l'extraordinaire attachement que les Français portent à leurs librairies indépendantes : alors que la fréquentation des salles de cinéma a chuté et que le chiffre d'affaires du spectacle vivant s'est effondré, contre toute attente, les librairies ont résisté, sans doute parce qu'elles matérialisent cette identité profondément littéraire de notre pays. En ces temps de divisions incessantes qui animent malheureusement notre vie politique, le parcours parlementaire de ce texte témoigne d'une forme d'union sacrée autour du livre et des librairies indépendantes. Les convergences de vues entre les deux chambres ont d'ailleurs conduit le Sénat à recourir à la procédure de législation en commission pour achever au plus vite l'examen du texte et rendre possible sa promulgation avant la fin de l'année. Avant cela, le Gouvernement, pour les mêmes raisons, avait engagé la procédure accélérée. Finalement, la commission de la culture du Sénat a adopté le texte à l'unanimité en seconde lecture. Demain, l'instauration d'un tarif minimal pour l'expédition de livres permettra un rééquilibrage de la concurrence dans le secteur du livre. la solidité financière de certains acteurs leur permettait jusqu'ici d'asseoir leur hégémonie grâce à deux avantages la décote de 5 % sur le prix des livres, autorisée par la loi Lang, et la gratuité des frais de port. Grâce au texte que nous votons aujourd'hui, ces derniers ne pourront plus contourner la loi de 2014 en proposant, par exemple, la livraison à 1 centime d'euro, au détriment des librairies indépendantes. Demain, les collectivités ou leurs groupements pourront attribuer des subventions aux petites librairies indépendantes. Cette disposition est une demande forte des élus locaux. Il sera ainsi possible de gérer au cas par cas les situations particulières qui adviennent sur chaque territoire et de financer le fonctionnement de ces petites librairies au-delà du seul investissement. Cette disposition permettra ainsi davantage de diversité culturelle et d'égalité d'accès à la culture. Demain, la réforme du contrat d'édition entre auteurs et éditeurs assurera une meilleure protection des auteurs dans le cadre des cessations d'activité des maisons d'édition. j'aimerais rappeler que l'instauration d'un tarif minimal de livraison pour les livres, qui a parfois pu faire débat parmi les acteurs de la filière, s'inscrit pleinement dans le prolongement de l'esprit de la loi sur le prix unique du livre, à laquelle les Français sont attachés. ans plus tard, cette loi aura permis de protéger la filière et de développer la lecture. Plus que jamais, elle a besoin aujourd'hui d'être complétée.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Le Sénat a adopté acteurs. L'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote sur la deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique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

monsieur le président de la commission, madame l'auteure et rapporteure, chère Sylvie Robert, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, nous arrivons donc, là aussi, au terme du processus législatif de la proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique.

Vous le savez, les bibliothèques constituent le premier équipement culturel public de proximité. Ces 16 500 établissements, en France, touchent un public très large, avec environ 12 millions d'usagers. Ce sont des lieux de culture à part entière où l'on s'informe, où l'on s'instruit, où l'on dialogue et où l'on s'enrichit. Ce texte arrive à point nommé et vient très justement compléter l'action engagée depuis 2017 en faveur des bibliothèques, sous l'impulsion du Président de la République, qui en avait fait un des axes forts de son programme. Ce quinquennat aura sans conteste permis de nombreuses avancées en la matière. Sur la base du diagnostic posé par Erik Orsenna et Noël Corbin en 2018, l'État et les collectivités territoriales ont renforcé leur collaboration pour étendre les horaires d'ouverture des bibliothèques, diversifier leur mission, accompagner la formation des professionnels. Grâce au plan Bibliothèques qui en est issu, l'État a accru les moyens alloués aux collectivités au travers de la dotation générale de décentralisation (DGD), des crédits importants du plan de relance pour 2021 et 2022, et d'une politique de contractualisation renforcée. Grâce à ces moyens nouveaux, une vraie dynamique est née et les résultats sont là. Entre 2016 et aujourd'hui, ce sont plus de 500 projets qui ont été soutenus dans toute la France. Les bibliothèques aidées ouvrent huit heures trente de plus par semaine par rapport à 2016. Cette politique offre ainsi la possibilité à près de 12,4 millions d'habitants, notamment dans les territoires les plus fragiles, d'accéder davantage à leur bibliothèque. Cette action en faveur de nos bibliothèques se concrétise aujourd'hui sur le plan législatif par l'initiative de cette proposition de loi qui va permettre demain, enfin, de consacrer le rôle essentiel des bibliothèques dans le code du patrimoine. Ce texte rappelle que les missions culturelles, éducatives, sociales et ludiques des bibliothèques s'inscrivent dans le respect des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions et de neutralité du service public. Les bibliothèques doivent demeurer des espaces de liberté, des lieux de respiration démocratique. Leurs professionnels doivent être protégés de la censure comme de toute pression politique, religieuse ou sociale. Leurs collections doivent refléter la diversité des opinions. Les bibliothèques doivent également rester accessibles à tous, librement et gratuitement. Il est important que la loi entérine un principe qui fait consensus et constitue l'une des conditions cardinales de leur succès. La loi accompagne, en outre, la montée en puissance des collaborations entre collectivités territoriales tout en respectant leur libre administration et en réaffirmant le rôle ô combien essentiel des bibliothèques départementales en soutien aux petites bibliothèques, notamment rurales. L'Assemblée nationale a enrichi le texte, et nous avons eu l'occasion d'évoquer en commission les avancées suivantes : la revente de livres par les bibliothèques de l'État et des collectivités territoriales à des entreprises de l'économie sociale et solidaire ; la disposition interdisant aux départements qui ont bénéficié du transfert par l'État d'une bibliothèque centrale de prêt de supprimer leur bibliothèque départementale ; ou encore l'ajout des notions d'accessibilité des personnes handicapées aux collections et aux services. Depuis le début de cette initiative législative, vous le savez, madame la rapporteure, j'ai exprimé le soutien sans faille du Gouvernement à ce texte. Le travail de qualité mené au Sénat puis à l'Assemblée nationale, en bonne intelligence et confiance avec le Gouvernement, permet aujourd'hui d'aboutir à un texte attendu, et qui rassemble tous les groupes. C'est là tout l'objectif de mon action au ministère de la culture depuis seize mois : rassembler et se rassembler pour faire vivre la culture.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je viens compléter le diptyque littéraire que nous offre cette matinée, après l'adoption définitive de la proposition de loi de Laure Darcos. La proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique, dont je suis à la fois l'auteure et la rapporteure, a été adoptée à l'unanimité au Sénat et à l'Assemblée nationale en première lecture, puis de nouveau à l'unanimité dans le cadre de la procédure de législation en commission le 23 novembre dernier.

matin. Comment ne pas s'en réjouir ? Comment ne pas y voir un formidable signal, une sorte de preuve d'amour-je le dis ! -adressée à l'ensemble des professionnels des bibliothèques, qui, je le sais, nous regardent nombreux en ce moment même ?

et, plus important, les valeurs et les missions, des bibliothèques. Il est difficile de croire que le premier équipement culturel du pays, avec 16 500 implantations, ne bénéficiait jusqu'à présent que de quelques dispositions législatives éparses et relativement floues dans le code du patrimoine.

Tous ont contribué à faire qu'aujourd'hui les bibliothèques disposent enfin d'un statut de référence qui leur est propre, fait d'exigence intellectuelle, de respect du pluralisme et de large ouverture pour tous. Je veux préciser aussi que ce texte s'adresse également à l'ensemble des élus locaux, qui ont cette belle responsabilité de gérer les bibliothèques. Ainsi, je suis particulièrement fière de voir aboutir à l'Assemblée nationale un combat qui me tenait à coeur, celui des bibliothèques départementales. Un nouvel article 9 A a en effet été introduit sur l'initiative du Gouvernement. Il précise que les départements ne peuvent pas supprimer, cesser d'entretenir ou de faire fonctionner les bibliothèques dont ils ont la charge.

J'espère donc que notre assemblée pourra ouvrir ce matin la voie à une promulgation rapide de ce texte, par un vote positif- je n'ose pas le souhaiter une nouvelle fois unanime, même si je l'espère très sincèrement ! Au terme de mon propos,

qui est à l'initiative de cette proposition de loi. C'est également l'occasion de rappeler l'importance de ce texte, très attendu, tant nous connaissons les vertus de la lecture et les bénéfices de ces lieux que sont les bibliothèques, si importantes à la vie culturelle de nos communes. Alors que des lois existent concernant les musées et les archives, jamais, jusqu'à ce jour, il n'y avait eu de loi-cadre sur les bibliothèques. C'est donc une première ! Pour la première fois, donc, ce texte donne une définition de ce qu'est une bibliothèque. La richesse que constituent les livres et la lecture est inestimable et je salue, à ce titre, le vote il y a quelques instants du texte de notre collègue Laure Darcos, qui permet de mettre en avant la filière professionnelle du livre et nos librairies. Lieux de rencontre, de partage, de savoir, d'apprentissage, de créativité, de liberté et d'émancipation, les bibliothèques répondent à de réelles attentes de nos concitoyens, qui sont attachés à ces lieux de vie pour petits et grands. 76 % des Français considèrent que les bibliothèques sont utiles à tous. Cette proposition de loi s'articule autour de trois grands principes qu'il était important de consacrer, afin de donner un cadre législatif clair, précis et ambitieux aux bibliothèques : la liberté d'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales, qui permet un accès sur place ou à distance ; la gratuité de l'accès à cet espace public et la gratuité de la consultation sur place ; et le pluralisme des collections, afin notamment d'éviter toute censure. inscrire les bibliothèques dans la loi permet également de reconnaître le rôle de l'ensemble des personnes qui y travaillent afin de les protéger : bibliothécaires, bénévoles et étudiants, dont le travail et l'engagement au service des autres sont à saluer. Les enjeux d'une bibliothèque en 2021 sont multiples : numériques, socioéconomiques, éducatifs, culturels. L'Assemblée nationale est venue compléter la liste des missions des bibliothèques territoriales. Il était utile de rappeler que les bibliothèques participent au développement de la lecture publique, à la réduction de l'illettrisme, à la diffusion et à la promotion du patrimoine linguistique, et à la coopération des organismes culturels, éducatifs, sociaux, mais également des établissements pénitentiaires. Aujourd'hui, on le voit au travers de leurs missions, les bibliothèques sont protéiformes et offrent des services qui s'adressent à toute la population. En évolution permanente, elles ont su se transformer pour relever ces défis sociaux, éducatifs et culturels. Elles ne sont plus seulement un lieu de savoir et d'études ; elles ont une vocation sociale et permettent la rencontre de toutes les générations et de tous les milieux socioprofessionnels. Par leur maillage territorial dense, les bibliothèques sont la première porte d'un égal accès pour tous à l'apprentissage et à la découverte de la lecture, avec tout ce que cela comprend. Ainsi, 70 % des communes de plus de 2 000 habitants ont une bibliothèque. Et nous voyons de plus en plus des projets de boîtes à livres émerger, notamment dans les rues des petites communes. Véritables services publics de proximité et parfois seul équipement culturel de la commune, les bibliothèques sont des lieux de vie auxquels les élus et nos concitoyens sont particulièrement attachés. En tant que sénatrice du Bas-Rhin, je tiens à prendre pour exemple la Bibliothèque d'Alsace, qui se caractérise par ses 700 000 ouvrages, 288 bibliothèques et 300 bénévoles investis. Son bon fonctionnement et l'engouement qu'elle suscite témoignent de la forte utilité des bibliothèques départementales. La proposition de loi que nous examinons a été adoptée à l'unanimité de notre assemblée le 9 juin dernier. Elle l'a également été le 6 octobre par nos collègues de l'Assemblée nationale, dont le travail a permis d'enrichir le texte. deux exemples : la possibilité donnée aux bibliothèques de l'État et aux collectivités de revendre les livres dont elles n'ont plus l'usage ; ou encore le fait que les départements ne pourront ni supprimer ni cesser d'entretenir les bibliothèques dont ils ont la charge. Je me réjouis réjouis que le processus législatif prenne fin, permettant ainsi à ce texte de voir le jour. C'est une fierté aujourd'hui et une belle reconnaissance pour tous les acteurs concernés, et je tiens de nouveau à remercier Sylvie Robert

c'est un plaisir de terminer l'année 2021 avec ces deux propositions de loi sur, d'une part, l'économie du livre et, d'autre part, les bibliothèques et le développement de la lecture publique. La lecture, les livres et les bibliothèques sont indispensables à la transmission des savoirs, mais aussi à l'ouverture sur le monde dont nous avons tant besoin. Je remercie de nouveau mes collègues Sylvie Robert et Laure Darcos, à l'initiative de ces textes. Grâce à vous, nous avons pu débattre au Sénat de ces sujets et obtenir l'unanimité sur ces deux propositions de loi. La proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique était très attendue par la profession. C'est grâce à leurs personnels que nos bibliothèques ont su innover, se réinventer, afin de sauvegarder cette richesse qu'est la lecture publique, sans oublier le rôle central de lien social qu'ils et elles maintiennent dans ces lieux. Le réseau de lecture publique s'est considérablement développé grâce en partie à la décentralisation. Dans le même temps, le cadre juridique dans lequel les bibliothèques territoriales s'inscrivent demeurait insuffisant. Cette loi apporte une réponse claire, adéquate et proportionnée à ce vide juridique. Pour cela, elle réaffirme trois grands principes essentiels : la liberté d'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales sur tout le territoire français la gratuité d'accès aux collections et documents présents dans les bibliothèques territoriales ; et, enfin, le pluralisme des collections afin de respecter les opinions de chacune et de chacun, et de réaffirmer la neutralité de nos services publics. Grâce à ces principes, nous pouvons avoir bon espoir que ce texte participe au développement de l'accès à la culture. En revanche, je regrette que le Gouvernement ait décidé de rendre obligatoire le passe sanitaire de 12 ans à 17 ans dans les bibliothèques, alors que dans le cadre scolaire le passe n'est pas demandé. Cette obligation risque d'accroître les inégalités d'accès à la culture. Après des mois de confinement avec l'école à la maison, il faudrait au contraire encourager les jeunes à se rendre dans les bibliothèques. L'Assemblée nationale a apporté à ce texte des ajouts intéressants, que je salue : sur le patrimoine linguistique, afin que les bibliothèques aient pour mission de participer à sa diffusion et à sa promotion, en écho à la proposition de loi sur les langues régionales adoptée en avril dernier sur l'accès aux personnes en situation de handicap, qui doit être facilité ; sur la réduction de l'illettrisme et l'illectronisme ; sur la coopération avec les organismes culturels éducatifs et sociaux et les établissements pénitentiaires enfin, sur l'impossibilité pour les départements de supprimer des bibliothèques ou de cesser de les entretenir. Je suis heureuse que les députés aient amendé l'article 12 dans le sens de ce qu'avec le groupe écologiste nous avions proposé en première lecture. Malgré la réserve du Sénat liée aux droits d'auteur, la mobilisation des bibliothécaires qui a suivi durant l'été a montré le non-sens de réduire les dons des documents uniquement aux associations loi 1901 sans possibilité de revente. L'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction qui permet aux bibliothèques de donner des livres dont elles n'ont plus l'usage à des fondations, à des associations philanthropiques ou à des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Celles-ci seront désormais autorisées à les revendre. Je le rappelle ici, cet article ne prenait pas du tout en compte les pratiques déjà existantes. Il aurait pu mettre en péril toute une économie du livre d'occasion, pour laquelle ces dons sont importants. Cela aurait malheureusement conduit à la destruction, à la mise au pilon, de trop nombreux livres. C'est avec enthousiasme que le groupe Écologiste-Solidarité et Territoires votera ce texte, qui répond aux enjeux et aux problématiques des bibliothèques et fait un pas vers une bibliothèque inclusive, gratuite et informée dans le choix de ses collections. La parole

Madame la présidente, madame la ministre de la culture et des archives, mes chers collègues, ce texte en apparence simple et technique porte une évolution majeure du statut culturel des bibliothèques. Il fonde la reconnaissance législative de la bibliothèque comme institution du service public de la culture, non seulement pour la promotion du livre et de la lecture, mais aussi comme relais territorial de proximité de l'action culturelle. Le nouvel article du code du patrimoine, créé par l'article 1 de la présente proposition de loi, donne enfin une âme à ce titre III, dont l'austérité toute notariale détonnait avec la place exceptionnelle que tiennent les bibliothèques dans notre imaginaire collectif des lieux du livre », mais aussi, et tellement, « des lieux du vivre », comme le disaient avec élégance Erik Orsenna et Noël Corbin dans leur rapport rendu le 20 février 2018. Notre collègue Sylvie Robert, auteure et rapporteure de cette proposition, dont je salue la qualité et la fulgurance du travail, fait sienne cette définition pour donner aux bibliothèques l'ambitieuse mission « de garantir l'égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs Vaste programme, aurait dit un général, et on peut d'ailleurs se demander si les bibliothèques ne vont pas finalement accueillir certaines des fonctions jadis dévolues, par son ministre de la culture André Malraux, aux maisons de la culture. Dans ce domaine, la proposition de loi va très loin puisqu'elle confère à cette mission générale toutes les garanties du service public, c'est-à-dire la neutralité, le pluralisme et l'interdiction de toutes les formes de censure idéologique, politique ou religieuse. Toutes ces règles sont elles-mêmes protégées par le principe de mutabilité du service public qui assurera leur pérennité, indépendamment de l'évolution des techniques, des procédés de lecture et des supports de l'information. Cette reconnaissance législative profite aussi et surtout aux personnels des bibliothèques et à leurs missions. C'est une évolution sociale considérable qui va sans doute imposer des adaptations de leur cadre d'emploi. En quelque sorte, les bibliothécaires rejoignent les rangs des hussards noirs de la République dans leur noble mission de « faire disparaître la dernière, la plus redoutable des inégalités qui viennent de la naissance, l'inégalité d'éducation », ainsi que le disait Jules Ferry en 1870. À l'heure de la prépondérance du numérique, de l'impérialisme abêtissant des plateformes et du mythe prométhéen de la capacité omnipotente de l'individu à se construire seul son capital culturel, il est réjouissant de constater la grande santé des bibliothèques. Partout où il en ouvre de nouvelles, elles sont rapidement victimes de leurs succès. Nous avons même observé combien la crise sanitaire a renforcé leur aptitude à offrir de nouveaux espaces d'échanges humains. Avec l'extension du télétravail, je ne doute pas que la bibliothèque va devenir pour beaucoup de salariés le dernier espace de socialité, un service public du vivre-ensemble. Il appartient maintenant aux collectivités de mettre en oeuvre les politiques publiques qui permettront aux bibliothèques de développer toutes leurs missions, dans un cadre juridique renouvelé. L'État doit les aider dans cette mutation ambitieuse. Ses responsabilités sont encore bien plus grandes s'agissant des bibliothèques dont il a la charge. Je pense aux bibliothèques d'école, mais aussi, et surtout, aux bibliothèques universitaires. La Cour des comptes a rendu, le 23 juillet dernier, un rapport accablant et alarmant sur la situation de ces dernières. Elle recommande au Gouvernement d'engager sans attendre des réformes de fond et des moyens budgétaires importants pour qu'elles puissent exercer leurs missions auprès d'étudiants qui sont dramatiquement privés de leur service. Les collectivités ne pourront continuer à accueillir celles et ceux qui ont renoncé à se rendre dans les bibliothèques de leur université. Il est urgent de mettre en oeuvre un plan de soutien de ces établissements, parce que, plus que tout autre établissement, les bibliothèques n'assurent pleinement leurs missions que dans un réseau homogène. En attendant l'ouverture de ce nouveau chantier- j'espère que vous allez vous en emparer, madame la rapporteure, avec la même réussite -, nous voterons sans réserve cette proposition de loi. La parole

on a parfois besoin que les choses nous manquent pour en réaliser la valeur. En effet, au plus fort de la pandémie, lorsque tous les lieux culturels avaient été contraints de fermer leurs portes, nombre de nos concitoyens ont ressenti ce manque.

de loi a pour mérite premier d'apporter une consécration aux bibliothèques, qui n'avaient jusqu'à présent pas de véritable texte-cadre. Ce sera bientôt chose faite. Je salue à ce titre la démarche et le travail très important mené depuis le mois de février dernier par notre collègue Sylvie Robert, auteure de la proposition de loi, en collaboration avec le président de notre commission et la ministre. Les bibliothèques sont aussi bien urbaines que rurales, aussi bien populaires que « bobos ». Elles ont cette capacité à se fondre dans tous les territoires, pour tous les publics ! Qu'elles soient municipales, intercommunales ou départementales, elles irriguent les territoires de culture, et c'est en cela qu'elles sont particulièrement importantes. Avec ce texte qui sera adopté tout à l'heure- j'en suis sûr -, certains principes fondamentaux seront gravés dans le marbre. Des principes particulièrement consensuels, tellement consensuels même que l'on est en droit de s'interroger sur l'opportunité de légiférer. Les principes inscrits dans le marbre à l'article 2 par exemple, à savoir le principe de gratuité d'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et de gratuité de la consultation, paraissent une évidence. En effet, quelle commune, quel élu local, prendrait la décision politiquement et socialement suicidaire de restreindre l'accès d'une bibliothèque ou de rendre la consultation des ouvrages payante sur place ? Je suis peut-être naïf de penser que jamais personne ne prendrait ce risque ! Alors peut-être qu'au final il vaut mieux que ce soit inscrit noir sur blanc. L'article 5 me paraît beaucoup plus important, surtout compte tenu du contexte actuel où la liberté d'expression est régulièrement menacée au nom de certaines idéologies. Peut-être que, grâce à cette loi, nous échapperons dans les bibliothèques françaises à des autodafés, comme cela s'est passé au Canada il y a quelques mois où 5 000 livres jugés stigmatisants ont été brûlés : on parlait là de bandes dessinées de Tintin et d'Astérix et Obélix ... Oui, la liberté d'expression c'est aussi accepter des ouvrages qui ne font pas l'unanimité, des ouvrages qui peuvent porter une vision dérangeante. J'approuve donc totalement cet article 5, mais m'interroge sur son articulation avec l'article 7 : celui-ci prévoit que les bibliothèques présentent leurs orientations documentaires à l'organe délibérant, présentation qui peut être suivie d'un vote. N'est-ce pas là le meilleur moyen de faire entrer de la politique ou de l'idéologie dans un domaine qui ne devrait pas en avoir ? Enfin, je mets l'accent sur l'article 8 qui consacre et offre une belle reconnaissance aux bibliothécaires. Car ce n'est peut-être pas le métier le plus connu, ni le plus reconnu, mais être bibliothécaire ne s'invente pas. Une bibliothèque vit par les livres et la documentation qu'elle peut offrir, mais pour tout cela il faut un chef d'orchestre, un maître d'oeuvre pour choisir les collections, guider, conseiller les lecteurs, leur donner le goût de la lecture et l'amour du livre. À l'heure où le livre ne fait plus toujours recette parmi la jeunesse, transmettre l'amour de la lecture et des livres est très important. Par ailleurs, alors que l'information n'a jamais été aussi facile à trouver, que la jeunesse est plus que jamais sujette aux, les bibliothécaires ont un rôle majeur à jouer dans cette éducation à l'information

c'est donc avec conviction et enthousiasme que le groupe Union Centriste votera en seconde lecture cette proposition de loi, qui grave dans le marbre certains principes de base, mais permet également de développer la lecture publique, un outil formidable d'émancipation et d'accès à la culture pour tous les Français. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le groupe du RDSE se réjouit du consensus qui a accompagné l'examen de ce texte sur les bibliothèques et le développement de la lecture publique. Les votes favorables, à l'unanimité, au sein de chacune des deux assemblées témoignent de l'intérêt que nous portons tous à nos bibliothèques locales. Cela a été rappelé, les bibliothèques prennent actuellement très peu de place au sein de notre corpus législatif. Par son adoption, la proposition de loi permettra de réparer cette anomalie et de briser ce silence surprenant au regard du rôle fondamental que jouent ces établissements sur l'ensemble du territoire. Grâce à l'initiative de notre collègue auteure et rapporteure Sylvie Robert, le code du patrimoine se verra ainsi enrichi d'une définition précise des missions des bibliothèques municipales, intercommunales et départementales, des missions qui dépassent depuis bien longtemps la seule conservation de livres et leur communication au public. « La marée montante des écrits, mais aussi la richesse des archives orales, le bouleversement et l'interdépendance des techniques de communication et d'information, la multiplication des supports que l'on dit éphémères parce qu'ils n'ont plus la pérennité du papier, tout cela oblige à redéfinir les perspectives et les moyens d'une mémoire organisée pour la postérité. C'est ainsi que François Mitterrand soulignait en 1988, dans l'un de ses discours, l'évolution à l'oeuvre concernant les bibliothèques et les archives. Il apparaît en effet important de soutenir constamment les bibliothèques face aux mutations qui les concernent. Les collectivités locales s'y emploient et vous l'avez rappelé, madame la ministre, l'État prend sa part, notamment au travers du plan Bibliothèques. C'est un effort qui doit être poursuivi, comme l'a suggéré le fameux rapport Orsenna-Corbin, notamment afin que ces établissements poursuivent du mieux possible leurs missions traditionnelles tout en amplifiant leurs fonctions plus récentes. Je pense en particulier à celle relativement nouvelle de réduction de l'illectronisme, d'ailleurs inscrite à l'article 1. Je profite de ce débat pour rappeler le travail engagé par le RDSE au travers de la mission d'information sur l'illectronisme conduite en 2020 par notre ancien collègue du groupe Raymond Vall. Son rapport évoquait les réticences de certains publics fragiles à aller vers les bibliothèques en raison de leur connotation culturelle et de la perception de ne pas être le public prioritaire. Il y a en effet encore trop d'usagers qui se sentent empêchés pour des raisons socioculturelles, ce qui peut atténuer en pratique la portée de « l'égal accès de tous à la culture Il est néanmoins important de rappeler ce principe à l'article 1, ainsi que celui de « libre » accès aux structures posé à l'article 2 du texte. Les bibliothèques ont fondamentalement une vocation humaniste. Le législateur doit y être attentif pour atteindre l'objectif beaucoup plus vaste d'inclusion sociale. L'accès au savoir est en effet au coeur du projet républicain. Nous devons l'honorer ; les collectivités locales l'ont bien compris lorsqu'elles déploient les bibliobus et leurs nombreuses initiatives autour de la lecture publique et du numérique. Dans cette perspective, les articles 9 et 9 A apporteront également leur pierre à l'édifice. Ils contribueront au maintien d'un maillage dense du territoire par les bibliothèques, une nécessité non seulement pour contribuer à la liberté d'accès que je viens d'évoquer, mais aussi pour garantir la diversité et le pluralisme de l'offre culturelle, principes que porte aussi la proposition de loi. Enfin, je n'oublie pas les bibliothécaires. Nous en connaissons de grands qui ont oeuvré dans le passé au sein de belles institutions : Marcel Proust à la Mazarine ou ici même au Sénat avec Leconte de Lisle et Anatole France. Ce sont des symboles de la culture française. Aujourd'hui, dans nos villes et villages, des milliers d'anonymes sont quant à eux les maîtres d'oeuvre de l'accès à cette culture. Ils méritent toute notre attention, tant la leur est toujours bienveillante à l'égard des usagers. C'est donc une bonne chose de les mentionner à l'article 8. Mes chers collègues, lieu de savoir, espace de travail, moment de rencontres intergénérationnelles, levier d'apprentissage de la lecture, mais aussi de l'usage du numérique, enjeu du dynamisme local

de voir clôturer ainsi ce matin une séquence autour du livre, que l'on peut considérer comme la principale porte d'entrée au monde qui nous entoure. La parole est à M. David Assouline, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Madame

la culture est un rempart contre tous les délires que certains distillent dans notre pays, le fracturant, misant souvent sur le manichéisme et la bêtise. Dans la culture, la question du livre a toujours été symbolique. Les fascistes ont commencé par brûler les livres.

On en recense plus de 16 000, ayant 12 millions d'usagers- la crise sanitaire n'a d'ailleurs pas empêché le nombre de ces derniers de croître, puisqu'ils étaient 250 000 de plus en 2020 par rapport à 2019. Cette adhésion aux bibliothèques s'explique notamment par la diversification de leurs activités et par l'évolution des usages. Le rapport Orsenna-Corbin révélait à ce titre que, si 40 % des Français fréquentent une bibliothèque au moins une fois par an, près de la moitié des usagers n'empruntent pas de livres. De sorte que les bibliothèques publiques deviennent progressivement des « tiers lieux », où l'on se rend pour avoir accès au wifi, boire un café, ou bien assister à des lectures publiques. L'absence de loi-cadre pour les bibliothèques pose aujourd'hui problème,

Cela rend évidemment nécessaire l'instauration d'un cadre législatif adapté qui, demain, permettra d'étudier d'autres questions, comme l'opportunité d'une inscription des bibliothèques départementales dans les compétences obligatoires des départements. Comme pour le texte précédent, cette proposition de loi fait l'objet d'un consensus assez inédit, que notre groupe salue : le Gouvernement a engagé la procédure accélérée et la commission de la culture a adopté le texte à l'unanimité en seconde lecture. montre combien le livre, dans notre pays, est capable de rassembler. Notre groupe votera naturellement en faveur de ce texte. La parole est à M.

nous examinons à présent la proposition de loi « Bibliothèques et développement de la culture publique », déposée par la sénatrice Sylvie Robert, dont je salue le travail et la ténacité en tant qu'auteure et rapporteure. Cette proposition de loi a été adoptée à l'unanimité par le Sénat le 9 juin dernier et par l'Assemblée nationale le 6 octobre. Madame la ministre, vous avez rappelé que, dans la lignée du rapport d'Erik Orsenna et de Noël Corbin, l'essentiel des dispositions de cette proposition de loi vient renforcer notre politique de la lecture publique, en dotant les bibliothèques des collectivités territoriales d'un cadre juridique à part entière. Les trois premiers articles forment la colonne vertébrale de cette politique. L'article 1 inscrit pour la première fois dans le code du patrimoine une définition claire des missions de ces bibliothèques qui maillent le territoire national. Relais Relais de culture autant que de lien social, les 16 500 lieux de lecture publique accueillent près de 27 millions de lecteurs chaque année, au bénéfice d'un public extrêmement diversifié. L'article 2 consacre pleinement le principe de liberté d'accès aux bibliothèques communales et intercommunales. Ce principe ne fait pas obstacle à l'instauration de jauges de fréquentation, indispensables à la sécurité sanitaire des lecteurs, en particulier en temps d'épidémie. L'article 3, essentiel, inscrit dans le marbre le principe de gratuité d'accès à ces mêmes lieux, ce qui n'est bien entendu pas incompatible avec les dispositifs d'abonnements payants mis en place par un grand nombre de ces bibliothèques. Nous devons différencier la consultation sur place des ouvrages et l'emprunt, lequel demande des garanties particulières pour assurer la pérennité des collections proposées. Au travers de ces principes de liberté d'accès et de gratuité, les bibliothèques contribuent à lutter contre l'illettrisme, qui touche encore deux millions de Français, mais aussi contre l'illectronisme- victimes de cette fracture numérique, 20 % des Français ne maîtrisent pas encore les principaux outils informatiques. Les bibliothèques sont de précieux relais de l'État dans les territoires- je pense en particulier aux et les bénévoles permettent d'animer la vie locale et d'accompagner des citoyens parfois très isolés socialement ou économiquement : aide aux démarches administratives, accueil des migrants, accompagnement des personnes âgées dépendantes, des détenus ou encore des personnes marginalisées Ces lieux de culture sont aussi des lieux d'intégration, participant pleinement à la restauration du lien social. En effet, l'accès à la culture en prison est l'une des clés de la réinsertion, si bien que deux tiers des bibliothèques situées dans de grandes villes ont des partenariats avec les prisons, les centres de semi-liberté et la protection judiciaire de la jeunesse. Si la lecture est le premier moteur de l'émancipation, c'est aussi un espace de transmission intergénérationnelle, propice aux partenariats entre école et associations de retraités. Les élus locaux et nos concitoyens y sont particulièrement attachés. Les principes consacrés par cette proposition de loi- la gratuité, la liberté d'accès, le pluralisme des collections et leur diversification -sont autant de principes fondamentaux constitutifs de l'ADN des bibliothèques locales. Les travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat ont permis de sécuriser et de préciser l'ensemble de ces dispositions. Cette convergence de vues a justifié le choix de recourir à la procédure de législation en commission pour cette nouvelle lecture au Sénat.

a associé en amont les professionnels du secteur, que ce soient les bibliothécaires, les libraires ou les éditeurs, puis, tout au long du parcours législatif, a veillé à associer le plus grand nombre autour des objectifs de ces propositions de loi, qui, je

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues,

groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.